jusqu'à 7 000 touristes par jour sur les sept kilomètres de long et trois kilomètres de large de la petite île de Porquerolles, dans le Var, 800 000 visiteurs par an dans les gorges du Verdon, 16 000 touristes par jour, l'été, sur la dune du Pilat, en Gironde, 49 navires commerciaux faisant des navettes sur la zone de la réserve de Scandola, en Corse, plus de 300 personnes par jour pour l'ascension du mont Blanc, en haute saison ; jusqu'à 30 000 touristes par jour sur le Mont-Saint-Michel au mois d'août ces chiffres hyperboliques décrivent une réalité, celle de nombreux sites protégés aujourd'hui partout en France. On parle « d'hyper-fréquentation » pour les cas extrêmes, sans atteindre forcément ces records, nombre d'espaces naturels sont aujourd'hui victimes d'un phénomène de saturation touristique, qui laisse les élus démunis face aux éventuels dommages qui en découlent pour la protection de l'environnement ou du caractère de ces sites. En tant qu'auteur de la proposition de loi, c'est à cette difficulté que j'ai tenté, modestement, de trouver une solution, aidé de nombreux juristes et spécialistes de ces questions, qui vivent, sur le terrain, ces difficultés. Nombre de collègues m'ont rejoint, puisque ce texte a été cosigné par des sénateurs issus de Les débats que nous avons eus en commission sont, de ce point de vue, révélateurs ; des marais salants de Loire-Atlantique, évoqués par notre collègue Christophe Priou, au massif du Mont-Blanc, dont nous a parlé Cyril Pellevat, en passant par les falaises d'Étretat, évoquées par Pascal Martin, et par la dune du Pilat, dont a fait état notre collègue Hervé Gillé tous ces exemples illustrent la difficulté de concilier une politique de tourisme durable avec la protection des sites naturels ou culturels patrimoniaux. Comme l'ont expliqué tous les acteurs que j'ai entendus, la forte fréquentation de ces sites tend à changer de nature et à se traduire par de nouveaux comportements. Le maire de Saint-Gervais-les-Bains, dans le massif du Mont-Blanc, évoquait

-pour la mettre sur les réseaux sociaux, mais qui, bien souvent, ne respectent pas les sites. Or ces nouveaux comportements peuvent avoir, sur l'environnement, des conséquences inattendues et importantes

L'objectif de la proposition de loi que nous nous apprêtons à examiner est de fournir aux élus un outil supplémentaire permettant de prévenir ces dommages. En effet, les outils qui existent aujourd'hui présentent certaines limites. Nous avons en France un principe fort, celui de l'accès libre et gratuit aux espaces naturels. Ce n'est pas du tout le cas partout dans le monde ; au au contraire, dans la plupart des pays, on paie pour entrer dans un site naturel. Cela dit, des outils de protection existent pour certains sites, en raison de leurs caractéristiques écologiques ou

À titre d'exemple, dans le coeur des parcs nationaux, le directeur de l'établissement public exerce un certain nombre de compétences attribuées au maire en matière de police. En outre, la charte de chaque parc, validée par un décret en Conseil d'État après consultation de l'ensemble des acteurs du territoire, peut également contribuer à la régulation de la fréquentation. Dans le cas des réserves naturelles nationales, l'acte de classement en réserve peut fermer et réglementer l'accès au site, ou définir un zonage plus restrictif. Il peut également réglementer les activités ou les manifestations sportives. En revanche, pour les sites classés, le classement ne permet pas de contrôler les usages ni les comportements inadaptés. Au-delà de ces outils juridiques, la plupart des acteurs mettent en avant l'importance des solutions pragmatiques, passant par l'aménagement du territoire dans le cadre de projets de territoire. À Étretat, par exemple, le réseau des grands sites de France a permis de mettre autour de la table tous les acteurs concernés, afin de trouver des solutions permettant de préserver le site du phénomène de l'hyper-fréquentation,

En effet, en tant que rapporteur, j'ai eu à coeur de travailler autant que possible avec neutralité et impartialité, d'écouter et d'entendre les critiques formulées par les différents acteurs que j'ai auditionnés. Nous avons procédé à une dizaine d'auditions, très intéressantes, très riches et très

m'ont alerté sur les difficultés que le dispositif initial pouvait soulever, notamment eu égard à son périmètre, qui était très large. J'avais été ambitieux, mais je ne le regrette pas ; j'avais pensé qu'il convenait de procéder à un élargissement, à la protection de l'environnement, encore un peu trop tôt pour cela. Toutefois, cette solution, qui mériterait d'être approfondie et travaillée, ne serait-ce que parce qu'elle reviendrait, selon moi, à tirer les conséquences des dispositions constitutionnelles de la Charte de l'environnement, était en réalité beaucoup plus large que l'objectif visé par le titre de la proposition de loi. Cet objectif consiste, je vous le rappelle, à permettre aux maires de réglementer l'hyper-fréquentation des zones touristiques, aux fins de préservation de l'environnement. Au cours des travaux, il m'a également été opportunément rappelé que la modification du pouvoir de police générale du pouvoir de police générale du maire conduisait également à lui confier une responsabilité nouvelle, et à l'exposer ainsi à d'éventuelles poursuites s'il ne s'en servait pas. Ce risque paraissait d'autant plus dommageable

alors que la plupart des polices spéciales de la nature sont exercées par l'État, une mauvaise interprétation de ces dispositions aurait pu laisser penser que les maires étaient désormais compétents, de manière générale, en matière de protection de l'environnement, et la délimitation précise de cette nouvelle compétence aurait été complexe, car « en creux » par rapport à l'ensemble des polices spéciales déjà attribuées, par le code de l'environnement, à d'autres autorités. Pour toutes ces raisons, la commission a recentré la proposition de loi sur une extension du pouvoir de police spéciale du maire, qui existe déjà en matière de circulation des véhicules motorisés- c'est l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales. Aujourd'hui, pour résumer, le maire ne peut qu'interdire les 4x4 sur certaines routes. La modification que nous allons, je l'espère, adopter, permettra à ce dernier, par un arrêté motivé, de réglementer également la circulation des personnes, par exemple, au sein d'espaces naturels hyper-fréquentés fragiles, dont les milieux seraient menacés. Cette solution présente l'avantage, d'une part, de ne pas conduire à des incompréhensions sur l'interprétation de ce nouveau pouvoir de police spéciale des maires, et, d'autre part, de limiter le risque de concurrence des polices spéciales. Je précise que cette solution a été travaillée en lien avec la commission des lois, dans la mesure où les pouvoirs du maire relèvent de son champ de compétence. Je tiens d'ailleurs à remercier tout particulièrement le président Bas, que j'ai pu consulter sur le texte ; il partageait la même analyse sur l'utilité d'un tel recentrage. Je conclurai en insistant sur le fait que ce nouveau pouvoir doit être vu comme un outil supplémentaire mis à la disposition des maires. La commission a prévu qu'un décret détermine les consultations nécessaires auprès des instances de gouvernance des espaces protégés, dans la mesure où les arrêtés ne seront efficaces que s'ils sont pris s'ils sont pris en lien avec les autres acteurs, dans le cadre d'un projet de territoire visant un aménagement et un tourisme durables. Voilà, mes chers collègues, en quelques mots, l'ambition de cette proposition,

Monsieur le président, monsieur le président de la commission, cher Hervé Maurey, monsieur le rapporteur, cher Jérôme Bignon, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi examinée aujourd'hui a pour objet de proposer un nouvel outil juridique pour trouver une solution aux différents problèmes que peut poser la sur-fréquentation de certains espaces naturels. Le développement de l'attrait et de l'intérêt de nos concitoyens pour les espaces naturels préservés et les paysages remarquables est grandissant. Il correspond à une attente, et même un besoin, de la part du public de pouvoir accéder à ces espaces et à ces sites. Nous ne pouvons que nous en féliciter ; cet engouement est aussi la récompense de la mobilisation de tous les acteurs qui travaillent au quotidien pour la politique de préservation des espaces naturels et paysagers.

France, deux territoires connaissant une fréquentation supérieure à 2 millions de visiteurs, Bonifacio, en Corse, et le massif de l'Esterel, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dès lors, le développement de la fréquentation de tous ces sites pose évidemment des difficultés d'un genre nouveau, auxquelles les outils permettant aux acteurs locaux d'agir ne sont pas totalement adaptés.

et au cumul des impacts : nuisances liées aux déchets, au bruit, au piétinement, aux dégradations des végétaux ou des équipements, à la difficulté de cohabitation entre les différents modes de loisirs.

Le cas du Mont-Blanc, ensuite, sur lequel nous avons été alertés par le maire de Saint-Gervais-les-Bains, permet d'illustrer les difficultés que peut causer la sur-fréquentation d'un site exceptionnel de haute montagne. Il y a en outre une particularité : le Mont-Blanc est protégé uniquement au titre de la réglementation relative aux sites classés, sites classés, qui ne permet pas de réguler, et encore moins d'interdire, une fréquentation excessive qui dégraderait ce site remarquable. S'il est possible, pour le maire ou le préfet, d'agir pour des raisons de sécurité, les autres nuisances et dégradations engendrées sur le site sont plus difficiles à encadrer.

Force est donc de constater que, malgré les outils existants, nous n'avons pas encore de réponse adéquate et que nous manquons de réactivité face aux situations qui se présentent.

Le Gouvernement est favorable à l'esprit général de ce texte, qui nécessitera probablement des ajustements au cours de la navette parlementaire, mais qui répond à une vraie urgence environnementale et politique. À ce titre, il paraît fondé que le maire puisse disposer, sur sa commune, de certaines prérogatives lui permettant d'agir, de façon motivée et proportionnée, pour contribuer à protéger ce patrimoine. Je souhaite toutefois porter à votre connaissance quelques points auxquels je suis attentive.

multipartite. Je suis donc attachée à ce que la mobilisation, par le maire, de cette nouvelle compétence puisse se faire en concertation et avec un avis de telles instances, lorsque celles-ci existent. Le problème de la sur-fréquentation des sites dépasse aussi le seul enjeu de la gestion des espaces naturels protégés, qui a vocation à permettre le bon état de conservation écologique ou de préservation paysagère du site.

l'hyper-fréquentation des sites naturels, culturels et patrimoniaux est un sujet préoccupant, qui évolue défavorablement. Le tourisme de masse est toujours en augmentation, en raison, souvent, de tropismes éphémères et de lieux considérés comme incontournables et immortalisés au moyen de selfies rapidement oubliés

Toutefois, la législation n'autorise pas un maire à réglementer ou limiter l'accès à certains sites dans la perspective de protéger l'environnement. En effet, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui précise les pouvoirs de police administrative générale du maire, fait reposer l'ordre public général sur trois piliers : la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. De ce fait, tout arrêté municipal initialement motivé par la volonté de protéger l'environnement ou le caractère d'un lieu ou d'un site est censuré, au motif qu'il n'entre pas dans ces champs.

En effet, dès les premières auditions, votre souhait d'accroître les pouvoirs de police générale du maire, partagé initialement par certains opérateurs territoriaux, a suscité des interrogations relatives aux conditions et au champ d'application Vous souhaitiez étendre ces pouvoirs de police à la préservation de l'environnement dans son ensemble, en autorisant le maire à intervenir pour prévenir toute forme d'atteinte à la protection des espèces animales ou végétales et de leurs habitats, et ce dans tous les sites bénéficiant d'un régime de protection en raison de leur dimension esthétique, écologique et culturelle. L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) a émis des réserves, et la poursuite de nos auditions nous a confortés dans cette analyse.

du code général des collectivités territoriales, qui met en place une police spéciale de la circulation dans les espaces naturels, au profit des maires. Cette disposition permettra de réglementer, et non pas seulement d'interdire, l'accès aux sites concernés, d'encadrer les pratiques touristiques et de supprimer la référence aux véhicules.

d'une manière plus globale, ce sujet suscite des questions sur la mise en oeuvre de la compétence tourisme ; cette compétence doit nécessairement s'inscrire dans un projet de territoire, cela a également été souligné, en organisant les subsidiarités, les processus de concertation et de coopération.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, alors que certains pays nordiques revendiquent un droit d'accès à la nature, cette proposition de loi vient rappeler trois éléments majeurs pour notre pays et nos concitoyens. D'une part, la France est le premier pays visité au monde. Avec près de 90 millions de touristes internationaux par an, les défis sont immenses et remettent naturellement nos politiques publiques en question, notamment dans un contexte de hausse exponentielle du tourisme mondial. D'autre part, les visiteurs et touristes recherchent plus d'authenticité et de connexion avec la nature. Enfin, de troisième part, nous avons, nous aussi, une tradition d'accès libre et gratuit à la nature, que nous tenons tous à voir perdurer. Le constat de Jérôme Bignon est sans appel : la saturation d'un certain nombre d'espaces protégés et son impact sur les écosystèmes interpellent les responsables de leur gestion et de leur préservation. cette semaine, le congrès des maires de France, la proposition de loi que nous examinons pose la question du rôle du maire dans la protection des sites naturels et culturels patrimoniaux, et de ses moyens d'action. La version initiale du texte prévoyait une nouvelle mission de police générale du maire, dédiée à la protection de l'environnement. J'y avais souscrit, en cosignant la proposition de loi avant même sa publication. J'y voyais un signal fort envoyé à nos élus, tout à fait en capacité de juger des mesures à prendre pour préserver un site d'intérêt sur leur territoire. au-delà de la consécration de la notion d'« ordre public écologique », en accord avec la conscience collective qui émerge dans notre société, un message d'espoir pour nos sites patrimoniaux, qui se voyaient octroyer un nouveau défenseur, au plus près du terrain. j'ai bien compris les risques que cette nouvelle mission faisait peser sur les maires. Si la décentralisation et la différenciation territoriale doivent être accentuées, il serait dommage de voir la responsabilité de la commune engagée en cas de dommages ou d'inaction, surtout dans un domaine aussi complexe que celui de l'environnement. du RDSE et moi-même souscrivons donc bien sûr à la rédaction adoptée en commission, qui permet au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, de réglementer et d'interdire la circulation des personnes dans certains secteurs. Nous vous proposerons toutefois deux amendements visant à l'enrichir. Le premier tend à rappeler qu'un site patrimonial s'étend rarement sur le périmètre d'une seule et unique commune, et que toutes les parties prenantes- collectivités, parc naturel, propriétaires -doivent être consultées dans le cadre d'un véritable projet de territoire. Le second a pour objet de rappeler que nous attendons depuis plus de trois ans la publication d'un décret, sur lequel j'ai interpellé, plusieurs fois, le Gouvernement, autorisant les agents assermentés des parcs naturels régionaux à rechercher et à constater les infractions en matière de protection du patrimoine naturel. Les gardes nature sont nos alliés en matière de protection de l'environnement ; ils connaissent le territoire comme leur poche et sont au plus près du terrain pour sanctionner les infractions. Nous devons pouvoir nous appuyer sur leur présence et leur expertise au quotidien. Cette proposition de loi a le mérite de rappeler l'importance de ces sites pour la biodiversité, au-delà de la beauté des paysages et du patrimoine culturel. Elle rappelle aussi que, malgré l'absence de régime général d'accès aux sites protégés, les collectivités font des efforts considérables pour canaliser les flux, avec des aménagements dédiés, et qu'il est sans doute nécessaire de voir émerger une politique touristique globale et cohérente de gestion des espaces naturels. L'équation est difficile à résoudre, entre la hausse de la fréquentation et la préservation des sites, elle-même indispensable à la poursuite de cette fréquentation. Plus le site est remarquable, plus il est fréquenté. À titre d'exemple, le département du Puy-de-Dôme, que je connais particulièrement, a la chance d'avoir fait inscrire, voilà un peu plus d'un an, la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'Unesco. Aujourd'hui, nous travaillons plus que jamais à l'émergence de politiques publiques permettant de faire rayonner ce site exceptionnel, de transmettre la connaissance par ce haut lieu tectonique et de ne pas le garder sous cloche, pour y faire prospérer le pastoralisme tout en le préservant du piétinement, des déchets et du comportement parfois peu civique des quelque 1,5 million de visiteurs qui s'y pressent déjà chaque année. des sites comme Venise, le Machu Picchu ou la baie de Maya en Thaïlande pourrait être durablement restreint, voire interdit, aux visiteurs. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour la France. Aussi, vous l'aurez compris, le groupe du RDSE votera en faveur de cette proposition de loi recentrée sur sa mission d'origine : réglementer l'hyper-fréquentation des sites touristiques pour les préserver durablement. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le tourisme, apparu en Europe au XIX siècle, est passé d'une pratique culturelle, réservée à une élite, à un phénomène de masse. Depuis les années 2000, ce secteur se développe de manière exponentielle partout dans le monde, et joue un rôle majeur dans l'économie mondiale. Le baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme évalue à plus de 1,4 milliard le nombre de touristes internationaux ayant voyagé en 2018, soit une augmentation de plus de 5 % en un an. Ce chiffre pourrait avoisiner les 2 milliards d'ici à 2030. Les dépenses des touristes ont aussi fortement augmenté. Les recettes engrangées par le tourisme international ont progressé de 4 % en 2018, s'élevant à 1 448 milliards de dollars ; ainsi, 4 milliards de dollars sont dépensés en moyenne chaque jour par les voyageurs. chaque jour par les voyageurs. La France est la première destination touristique au monde, avec quasiment 90 millions de visiteurs étrangers attirés en 2018. L'Hexagone bat son propre record de fréquentation et s'approche du cap des 100 millions de visiteurs, qui pourrait être dépassé en 2020. Il est indéniable que le tourisme est un secteur vital de l'économie française, au vu de ses retombées financières. Si ces retombées sont vitales pour notre pays, l'hyper-fréquentation- le « sur-tourisme » -a des conséquences néfastes, tant pour l'environnement que pour les habitants des régions concernées. Nous sommes nombreux à avoir ainsi à l'esprit l'image du paquebot de treize étages qui a heurté un quai et un bateau en voulant s'amarrer en juin 2019 à Venise. Le pire a été évité, mais, au-delà du danger physique que ces accidents peuvent occasionner pour les touristes, ces géants des mers contribuent à l'érosion des fondations de la ville, alors que celle-ci et sa lagune sont inscrites au patrimoine mondial Le gouvernement italien a réagi en interdisant l'accès du centre historique aux paquebots géants. Entre la manne financière substantielle et la véritable menace pour la survie de la ville, il semble que la raison l'ait emporté. En France, nous ne sommes pas en reste : habitants excédés, sites naturels ravagés ou pollués, villages muséifiés ... Les dégâts du tourisme de masse sont légion. Je ne reprendrai qu'un seul des chiffres essentiels

Face à cette situation, la préfecture de Haute-Savoie a mis en place une série de mesures de régulation de l'accès au mont Blanc assorties de sanctions pénales et administratives particulièrement dissuasives. dissuasives. Face à la détérioration continue de la situation, les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités en protégeant un site classé et en assurant mieux la sécurité des visiteurs. Plus généralement, face à cette pression touristique, les autorités locales adoptent des mesures pour protéger villes et populations. Certaines villes françaises voient leur population se multiplier avec la venue des touristes, créant ainsi d'importants déséquilibres au niveau local : rues et transports surchargés, nuisances sonores, plages bondées ... Les commerces de proximité cèdent la place à des bars et à des boutiques de souvenirs. La prolifération d'hôtels et d'hébergements touristiques engendre une pénurie de logements pour les habitants et une hausse des prix de l'immobilier. Certains lieux ne sont pas adaptés pour recevoir un trop grand nombre de voyageurs et manquent d'infrastructures.

Plus généralement, le sur-tourisme accentue le phénomène de gentrification, le départ des classes populaires des centres-villes au profit d'une classe sociale plus aisée. Face à l'augmentation du coût de la vie, les habitants sont contraints de se loger ailleurs et les quartiers se vident progressivement de leurs habitants. Le sur-tourisme exerce inévitablement des pressions sur l'environnement, avec une surconsommation des ressources naturelles, une part plus importante de déchets dans la nature, une pollution accrue de l'eau et des sols qui nuit à la biodiversité, la destruction des écosystèmes, la disparition de la biodiversité. Sur ce dernier point, un phénomène inquiétant jour : des lieux préservés, encore inconnus voilà quelques années, et popularisés par les réseaux sociaux sont aujourd'hui gravement menacés par l'afflux massif de touristes. En France, il existe un principe primordial de libre accès et de gratuité des espaces naturels. Toutefois, plusieurs outils permettent de protéger certains sites eu égard à leurs caractéristiques environnementales ou culturelles patrimoniales. Ainsi, un grand nombre de polices spéciales de la nature vise à assurer la préservation des espaces naturels et des espèces de la faune et de la flore sauvages. Par ailleurs, la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a instauré une taxe destinée à faire participer les passagers du transport public maritime à la protection d'espaces protégés, qu'ils y débarquent ou non. En outre, En outre, plusieurs solutions d'aménagement du territoire, concertées au niveau local, visent à remédier aux problèmes liés à la sur-fréquentation des sites et espaces naturels. Cependant, il n'existe pas de régime général d'accès aux espaces naturels et aux sites bénéficiant d'un régime de protection. cela a déjà souligné, notre commission a modifié la proposition de loi initiale portée par Jérôme Bignon, en recentrant le dispositif sur l'extension du pouvoir de police spéciale de la circulation des véhicules motorisés. Le maire pourra ainsi réglementer, et non plus seulement interdire, l'accès et la circulation des personnes, et non plus des seuls véhicules motorisés, sur certaines voies ou dans certains secteurs, dès lors que cet accès serait de nature à y compromettre la préservation de l'environnement. Le maire disposera ainsi d'un outil supplémentaire pour préserver des sites bénéficiant d'une protection pour des raisons écologiques ou culturelles, dont le caractère serait menacé par une hyper-fréquentation touristique. Comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises, il ne s'agit que d'un premier pas

en est. Le tourisme est une activité de premier plan pour l'emploi et l'économie de la France et de ses territoires. Si les retombées économiques sont vitales pour notre pays, la préservation de notre patrimoine culturel et environnemental l'est tout autant. Il s'agit aujourd'hui de stopper les conséquences mortifères du tourisme de masse et de favoriser le développement d'un tourisme éco-responsable, en donnant aux maires la possibilité de réguler l'activité touristique pour qu'elle soit plus raisonnable et mieux encadrée.

nous ne pouvons que souscrire à cette proposition de loi dont je tiens à remercier l'auteur et rapporteur, Jérôme Bignon. Ce texte vise à mieux protéger les sites d'un tourisme de masse incompatible avec la protection de la nature et de la biodiversité,

d'une véritable prise de conscience des enjeux environnementaux. Le principe de police administrative générale donnée au maire ne permet pas actuellement, selon une jurisprudence constante, et malgré la référence à la lutte contre les pollutions de toute nature, de traiter de l'hyper-fréquentation des sites et du tourisme de masse. Ainsi, l'ordre public recouvre aujourd'hui uniquement le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Faire évoluer la notion même d'ordre public nous semblait une démarche innovante et porteuse de sens, une évolution d'autant plus souhaitable que la notion d'ordre public, par nature mouvante, doit pouvoir s'adapter aux nouveaux besoins. Dans ce sens, et alors que nous avons intégré la Charte de l'environnement au bloc de constitutionnalité, bousculer la définition de l'ordre public nous semblait légitime, voire même souhaitable. Cependant, nous entendons vos arguments sur le caractère trop général d'un « ordre public écologique » aux contours trop vastes qui entraînerait des risques d'interprétation juridique hasardeuse et, donc, une incertitude pour les maires chargés d'une compétence en contradiction avec des polices de l'environnement supportées par d'autres acteurs.

cette police, qui ne traitait initialement que de la circulation des véhicules, à la notion de fréquentation générale. Au final, le résultat sera le même et c'est bien cela qui compte. Nous sommes donc d'accord avec cette évolution législative, malgré quelques questionnements d'ordre plus général.

remarquables et des merveilles de ce monde. Au Bhoutan, par exemple, le nombre de visiteurs étrangers est limité par une taxe de séjour quotidienne très importante. Nous portons, pour notre part, la conviction que la régulation de fréquentation ne peut se faire en instaurant un droit d'entrée payant, ce qui reviendrait à interdire l'accès de ces sites Le principe de gratuité d'accès aux espaces naturels doit être maintenu. Par contre, la régulation par des inscriptions ou par l'interdiction intermittente d'accès permettant de limiter le nombre de présents nous apparaît opportune. opportune. Une politique de prévention sur les sites pourrait également être mise en oeuvre pour favoriser un tourisme responsable et durable, et accompagner ainsi les élus dans leur démarche. Nous pourrions d'ailleurs intégrer cette mission à l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui va entrer en fonction très bientôt. Pour autant, s'il est légitime de donner aux élus les moyens de préserver leur territoire, encore faut-il qu'ils puissent également financer les remises en état et la préservation des sites sur le long terme, notamment dans le cadre de leur politique d'aménagement. Or les dotations aux collectivités sont limitées et la préservation de l'environnement est souvent le parent pauvre des politiques locales. Enfin, l'État ne peut se désintéresser de la question de la protection de la biodiversité des sites remarquables, qui font parfois l'objet d'une protection particulière au titre du code de l'environnement.

43 pour le seul Office français de la biodiversité, en parfaite contradiction avec l'objectif affiché de faire de la préservation et de la reconquête de la biodiversité une priorité de l'action en matière environnementale. L'État doit prendre sa part de responsabilité. Pour finir, nous pensons qu'il convient, en parallèle de cette régulation et de ce nouveau pouvoir octroyé aux maires, d'engager une réflexion sur le tourisme de masse et le modèle économique qu'il sous-tend en favorisant un éco-tourisme plus respectueux de notre environnement dans une vision de long terme, soutenable pour l'humanité. Nous devons donc changer de modèle de développement et de tourisme, par exemple en pénalisant plus fortement les mobilités polluantes, en régulant les capacités de tourisme sur certains territoires et en limitant drastiquement l'artificialisation des sols qui défigure nos côtes, nos montagnes et les espaces les plus fréquentés.

madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'homme cueilleur-chasseur a toujours évolué dans la nature. Son territoire était restreint et respecté, car il y allait de sa survie. Aujourd'hui, l'homme hyper-consommateur veut aller partout, le plus rapidement possible, en oubliant parfois le respect de l'endroit et, malheureusement, en laissant chaque fois une trace de son passage. Pourtant, les territoires naturels sont fragiles, les sites abritent des écosystèmes rares et une biodiversité riche. Dans beaucoup de cas, la réglementation, voire l'interdiction de l'accès au public, est indispensable sur les sites sensibles.

et comprendre ces derniers aide à mieux les protéger tout en permettant au plus grand nombre de découvrir les richesses de la nature. Parce que certains sites naturels doivent être protégés, il nous faut un arsenal juridique qui nous autorise à le faire.

a constaté que le dispositif de régulation de la fréquentation des lieux menacés était insuffisant. Nous devons protéger durablement les milieux naturels, en concertation avec les acteurs locaux. Merci à lui de proposer ce texte. Dans sa première mouture, la proposition de loi n'était pas satisfaisante en ce qu'elle conférait au maire un pouvoir général de police environnementale- donc trop large -qu'il aurait été bien en peine d'exercer et qui l'aurait exposé à d'infinies poursuites. Il faut des mesures adaptées. Le pouvoir de police du maire est une condition indispensable à la préservation des milieux d'intérêt écologique et à la protection des sites. Heureusement, Jérôme Bignon a modifié son texte avec pertinence en élargissant simplement le pouvoir de police spéciale de la circulation du maire.

s'agit donc d'un bon texte, que nous voterons. En complément, je pense que l'Office français de la biodiversité, ce nouvel opérateur pour protéger et restaurer la biodiversité et dont les missions sont de simplifier l'organisation par le rapprochement des expertises, coordonner pour renforcer l'efficacité des politiques publiques et de renforcer l'action territoriale pour garantir un partage équilibré des usages et des espaces naturels,

Nous avions, à l'époque, établi des dossiers d'indemnisation, la saison touristique 2000 ayant été catastrophique. Nous nous étions aperçus en Loire-Atlantique, en Vendée, en Pays de la Loire que le tourisme arrivait bien loin devant toutes les économies

les dernières données de l'Organisation mondiale du tourisme sont claires : le tourisme n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Il représente environ 10 % du PIB mondial. Les prévisions pour les années futures confirment cette tendance. La France est la destination la plus prisée, avec près de 90 millions de touristes pour l'année 2017. L'arrivée de touristes dans notre pays est une excellente nouvelle pour le rayonnement de sa culture et la beauté de nos territoires. Toutefois, cela nous oblige à nous poser la question des conséquences de ce phénomène, notamment en cas de fréquentation massive. Je tiens donc à saluer le travail pertinent et neutre entrepris par le rapporteur, notre collègue Jérôme Bignon, ainsi que la justesse du calendrier. Les élections municipales sont dans quelques mois- autant dire demain -et les propositions des maires et des candidats sur le tourisme seront primordiales dans beaucoup de nos territoires. Nous sommes face à l'inévitable confrontation entre la fréquentation souhaitée de nos sites touristiques et culturels et leur préservation. La fréquentation touristique est souvent une chance, à la fois pour nos territoires, en termes de croissance économique, mais aussi pour les visiteurs. Ce tourisme est un moyen de transmission, d'éducation, de sensibilisation aux enjeux de préservation et de découverte de notre histoire. Nous voyons de nouvelles formes de tourismes apparaître avec une conscience forte de l'impact de cette activité sur les sites touristiques- mais pas seulement. Les selfies à la chaîne et le besoin désormais vital de poster sur les réseaux sociaux chaque instant instant insignifiant de nos vies ont également entraîné un tourisme de consommation. Tout comme on ne regarde plus une oeuvre dans un musée pour s'assurer seulement d'en avoir capté l'essence en photo pour la partager,

Ces nouvelles pratiques n'ont pas toujours un effet négatif sur le tourisme et ont permis de faire découvrir au grand public des sites hors normes. L'attractivité a aussi permis d'alerter sur des sites en danger que l'humanité ne peut se permettre de voir disparaître. Cependant, elles ont aussi eu des effets néfastes sur certains lieux aux prises avec une hyper-fréquentation qui n'avait jusque-là pas été envisagée. Les impacts sont majoritairement environnementaux. La fréquentation massive peut entraîner une saturation des sites avec des conséquences sur la biodiversité, même sur la sécurité. Les sites peuvent être abîmés ou fragilisés par le passage trop fréquent de véhicules ou de personnes. Les conséquences sont parfois dommageables pour le tourisme lui-même. La question des pollutions diverses est également un enjeu. Les déchets sont un exemple parmi tant d'autres. La pollution sonore et la qualité de l'air peuvent ainsi avoir un impact et fragiliser tout un écosystème. De manière générale, les touristes, et donc les citoyens, doivent se responsabiliser quant à leurs gestes et à leurs actions afin de pouvoir profiter de manière durable des endroits qu'ils visitent et les transmettre aux générations suivantes. Dans le monde entier, des mesures ont été prises. Les cas sont assez nombreux. Je n'en citerai qu'un, celui de l'Indonésie, qui réfléchit à restreindre l'accès, de manière temporaire, à l'île de Komodo, refuge de ses célèbres dragons menacés, entre autres, par la venue de milliers de touristes chaque semaine. ce phénomène d'hyper-fréquentation reste ciblé sur certains lieux qui ont acquis une notoriété incontestable comme le Mont-Saint-Michel, le Mont-Blanc ou encore les gorges du Verdon. Mais d'autres lieux en font également les frais en période de grande affluence. Des outils déjà existants sont utilisés par les responsables locaux, comme l'a très justement mis en exergue Jérôme Bignon dans son rapport. De meilleurs aménagements de sites pouvant accueillir plus de personnes pouvant accueillir plus de personnes en toute sécurité sont réalisés. À l'extérieur des sites également, avec la construction de parkings pour éviter l'usage de la voiture, ou des places de stationnement encadrées pour réguler la fréquentation. Dans certains lieux, des éco-gardes sont présents pour s'assurer du respect des règles et alerter sur les bons gestes. Les maires particulièrement ont un panel de solutions à leur disposition avec des pouvoirs en matière environnementale, qu'il s'agisse de pollution ou de prévention. Ces outils fonctionnent et sont reconnus comme efficaces. La proposition qui nous est faite vient compléter le dispositif déjà existant et le parfaire. Elle crée une nouvelle police spéciale à l'endroit des maires qui pourront désormais réguler l'accès à certains sites ou zones de site.

Cependant, la flèche pourra être retenue avant d'atteindre sa cible, car l'arrêté motivé devant être délivré suppose la discussion avec des acteurs locaux. Cela renforcera certainement le pouvoir de la décision et sa justesse. Ainsi, la fréquentation massive de nos sites naturels et culturels patrimoniaux est un double enjeu. De préservation, certes. Mais rappelons-nous que beaucoup de nos territoires espèrent une forte attractivité pour le partage de la beauté de leurs sites, pour le rayonnement de leur histoire et de leurs spécificités. C'est ce que nous espérons tous. La France a des atouts formidables. Chaque fois que cela sera nécessaire, une boîte à outils renforcée sera disponible afin de préserver ces richesses. De leur côté, nos concitoyens, et les citoyens du monde, doivent aussi se sentir concernés et responsables afin qu'ensemble nous préservions notre bien commun et les témoignages de notre patrimoine.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les connaisseurs du patrimoine savent bien que l'hyper-fréquentation des sites culturels et naturels peut être un véritable problème.

du phénomène. Le cas de Venise est connu et emblématique. Lors d'un déplacement effectué en octobre 2016, notre commission de la culture a pu constater sur place la menace que fait peser le tourisme de masse exode des habitants, surexploitation inappropriée des ressources, dégradation continue du système écologique et culturel de Venise et de sa lagune. À tel point que, le 2 octobre dernier, le comité du patrimoine mondial de l'Unesco a annoncé envisager d'inscrire Venise sur la liste du patrimoine mondial en péril si des progrès significatifs n'étaient pas faits pour en assurer la conservation. Et Venise n'est pas un cas isolé. Le phénomène ne peut que s'emballer dans les années qui viennent. Selon l'Organisation internationale du tourisme,

La présente proposition de loi s'inscrit donc dans la droite ligne de cette prise de conscience. Je remercie vraiment notre collègue Jérôme Bignon d'en avoir eu l'initiative. Ce texte entend donner aux maires les moyens juridiques de lutter contre l'hyper-fréquentation des sites naturels et culturels. Lier sites naturels et culturels est en parfaite adéquation, je tiens à le dire, avec la réflexion que nous avons menée, ici, au Sénat lors des débats sur la loi l'architecture et au patrimoine, en créant les sites patrimoniaux remarquables. Par ailleurs, je le rappelle, le Comité national des biens français est placé sous la double tutelle du ministère de la culture et du ministère de l'environnement.

je tiens à féliciter notre collègue Jérôme Bignon, avec qui je partage de nombreuses actions, d'avoir pris l'initiative de cette proposition de loi et d'avoir travaillé sur la protection de notre cadre de vie et l'enrichissement des moyens mis à disposition des maires dans l'exercice de leurs fonctions. de leurs fonctions. Ce texte vient mettre en lumière les nouveaux défis que nous devons relever. Trois d'entre eux me semblent particulièrement prioritaires : répondre intelligemment et concrètement à l'explosion mondiale du tourisme,

Le sujet est vaste, aussi riche que la réflexion qui s'impose, mais la rédaction de cette proposition de loi vient contribuer de façon positive aux actions engagées. Incontestablement, nous devons nous réjouir de l'attractivité dont bénéficie notre pays : nous recevons de plus en plus de touristes. L'Organisation mondiale du tourisme estime que, d'ici à 2030, 4 millions de touristes s'ajouteront au 1,4 milliard de personnes qui voyagent déjà. À l'heure où la concurrence mondiale pour capter la venue de touristes est forte, la hausse de la fréquentation touristique en France est le signe d'une réelle vitalité et la conséquence de politiques touristiques efficaces. efficaces. Reste que cela ne nous autorise pas à faire n'importe quoi, n'importe comment. Pour de nombreuses destinations, gérer cet essor représente un défi important.

les moyens légaux mis à la disposition des élus pour encadrer cet afflux de touristes ne sont pas adaptés. Parfois, des actions menées pour la protection de l'environnement peuvent provoquer le contraire de ce que nous voulions.

J'approuve le texte adopté par la commission, lequel, en recentrant plus précisément les dispositifs à faire évoluer, témoigne de pragmatisme.

Il était difficilement envisageable d'exposer les maires à des responsabilités nouvelles. Ils en ont déjà bien assez ! Cela les aurait potentiellement exposés à des poursuites pour inaction fautive, alors même qu'ils ne disposent pas, le plus souvent, des moyens techniques, juridiques et humains appropriés. En outre, alors que la plupart des polices spéciales de la nature sont exercées par l'État, une mauvaise interprétation de ces dispositions aurait pu laisser penser que les maires sont désormais compétents de manière générale en matière de protection de l'environnement. L'accent a donc été mis sur la cohérence entre les différents dispositifs. Je crois particulièrement à l'efficacité de cette démarche. Néanmoins, une telle initiative en appelle bien d'autres. Notre gestion globale du tourisme évolue-t-elle assez vite face à un risque climatique qui nous alerte de plus en plus, alors que nos concitoyens aspirent à retrouver des liens plus vrais avec la nature ? Rien n'est moins sûr ! Les qualités naturelles et paysagères restent en effet un facteur essentiel de l'attractivité des territoires de par le monde. Le tourisme, par son caractère transversal, en appelle à une réponse globale, avec une véritable coordination des outils et un partage des responsabilités.

en forêt de Fontainebleau pour profiter de ses charmes et pour le plaisir de gravir quelques-uns des plus beaux blocs de grès de la planète. Il y avait là quelques « bleausards », les habitués de cette forêt,

de loi portant diverses mesures tendant à réguler « l'hyper-fréquentation » dans les sites naturels et culturels patrimoniaux constitue l'autre bout de l'omelette, si vous me passez cette expression chère au Premier ministre. Le Sénat, dans sa grande sagesse, souhaite préserver la possibilité de fouler les plus beaux sites naturels, mais il veut aussi préserver leur pérennité et, donc, éviter l'hyper-fréquentation si bien décrite dans le rapport de Jérôme Bignon. Sont notamment concernés la baie de Somme avec ses embouteillages sur plusieurs sorties d'autoroute, Port-Cros et ses nombreux allers-retours de bateaux ou encore le Mont-Blanc et ses faux guides. Les dérives en matière d'accès à certains de nos plus beaux sites naturels sont nombreuses ! Ce texte évite les pièges que beaucoup ont décelés durant l'examen du projet de loi Engagement et proximité, à savoir donner des pouvoirs de police aux maires, ce qui les mettrait en première ligne sans leur donner les moyens d'exercer leur compétence. En prévoyant d'élargir la portée de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, qui met en place une police spéciale de la circulation dans les espaces naturels au profit des maires, il aboutit à une solution pragmatique. Avec mes collègues du groupe socialiste, nous présenterons un amendement qui s'inscrit dans le périmètre de cette proposition de loi. Il vise à apporter une réponse ferme aux inconscients égoïstes qui seraient tentés de renouveler l'atterrissage sauvage accompli il y a quelques mois au sommet du mont Blanc, pour une dépose peu compatible avec les usages et le respect de la montagne. J'avais déposé une proposition de loi sur ce thème et recueilli nombre de réactions positives. J'ai cependant retravaillé le texte en échangeant avec le Gouvernement, afin d'éviter que les pilotes de bonne foi et soucieux de l'environnement ne pâtissent de mes suggestions. Nous aurons l'occasion tout à l'heure d'évoquer ce sujet plus en détail. Nous sommes tous sensibles à ces questions sur lesquelles nous pouvons nous retrouver en laissant de côté les étiquettes politiques. Le Président de la République s'est exprimé sur le Mont-Blanc ; on imagine qu'il est également sensible à la question de la baie de Somme, qui vous est chère, monsieur Bignon. Nous espérons donc que le Gouvernement sera attentif à nos débats. D'ici là, j'espère que vous me pardonnerez de contribuer à l'hyper-fréquentation de l'hémicycle ce matin, bien que je sois membre de la commission des lois, pour présenter un amendement qui ne concerne même pas mon département. Mais je crois que votre texte intéresse largement et que le Mont-Blanc mobilise tous les Français,

: La parole est à M. Éric Gold. Le présent amendement vise à ce que le pouvoir de police spéciale du maire réglementant l'accès aux espaces protégés s'exerce dans le cadre d'un projet de territoire, en précisant que le décret en Conseil d'État prévoit les modalités de consultation des parties prenantes locales

est ainsi libellé : La parole est à M. Jérôme Durain. L'atterrissage d'un avion de tourisme au sommet du mont Blanc le 18 juin dernier a mis en lumière le caractère lacunaire de notre arsenal législatif pour lutter contre ce type de comportement, qui contrevient aux usages en vigueur en montagne et transgresse les lois en matière de protection de l'environnement. En Haute-Savoie et au-delà, ce comportement déplorable a légitimement choqué celles et ceux qui aiment la montagne et souhaitent que son environnement soit préservé. Certes, l'article L. 363-1 prévoit déjà que, dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont interdites, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l'autorité administrative. Toutefois, à défaut de sanctions dans les textes, cette interdiction ne peut aujourd'hui être mise en oeuvre. Le pilote incriminé le 18 juin dernier n'a écopé

sont inquiétés des conséquences possibles sur les aérodromes de Saint-Rémy-de-Maurienne et Sollières et sur les pratiques responsables d'aviation de montagne. J'ai été heureux d'échanger avec le cabinet de Mme la secrétaire pour parfaire cet amendement. Selon moi, sa rédaction permet désormais d'éviter toute conséquence néfaste pour les pilotes qui respectent les règles et de rester dissuasif pour ceux qui seraient tentés de renouveler le triste exploit du mois de juin. Le Président de la République a eu l'occasion d'en faire part, est conscient des enjeux de préservation du Mont-Blanc, qui dépassent la seule question des atterrissages sauvages. J'espère que le présent amendement aidera les élus de ce département, qui n'est pas le mien, à préserver notre patrimoine naturel national. Quel est l'avis de la Quel est l'avis de la commission ? À la suite de divers incidents, notamment l'atterrissage d'un avion de tourisme au sommet du mont Blanc en juin, cet amendement vise à renforcer les dispositions prévues par notre droit sur le sujet. à interdire l'atterrissage et la dépose de personnes par aéronef motorisé à des fins de loisirs, en assortissant cette interdiction d'un régime de sanctions pénales lourdes, puisqu'il s'agit d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende et de six mois d'emprisonnement et de 75 000 à interdire la dépose de personnes par aéronef non motorisé, mais sans la soumettre au régime de sanctions pénales prévues pour le premier cas. En effet, il paraîtrait disproportionné de sanctionner pénalement quelqu'un qui atterrirait en deltaplane, par exemple. Ce sujet rejoint tout à fait les préoccupations de la proposition de loi que nous examinons, laquelle tend à compléter la boîte à outils permettant de faire face aux nouvelles habitudes touristiques auxquelles sont confrontés de nombreux sites naturels aujourd'hui

un régime de sanctions et de mieux encadrer l'atterrissage d'aéronefs dans des zones sensibles, sans pénaliser les acteurs de bonne foi et avec le bon régime juridique. Je veux saluer le travail très constructif mené

Cet amendement vise à appeler l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'un décret, promis depuis plusieurs années, visant à l'assermentation des gardes nature au sein des parcs régionaux. En juin 2018, en réponse à une question posée, le ministre de la transition écologique et solidaire avait promis ce décret d'application l'année 2018. Lors de l'examen du projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, le Gouvernement avait annoncé sa publication pour l'automne 2019. Or ce décret n'est toujours pas paru, laissant les gardes nature démunis de leurs possibilités de constater des infractions, au détriment de la protection de notre patrimoine naturel.

Il me semble donc que je pourrai tenir l'engagement que j'avais pris lors de l'examen de la loi portant création de l'Office français de la biodiversité de sortir ce décret d'ici à la fin de l'année, peut-être même techniquement à l'automne 2019, puisque, l'hiver arrivant le 20 décembre,

Merci